avant la disparition de plus en plus probable du verrou de Bercy et la banalisation de la procédure pénale en matière de délinquance financière, notamment de fraude fiscale. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, familièrement dénommée « plaider-coupable », a été instituée en droit français par la loi du 9 mars 2004 Dans le cadre de cette procédure, la personne qui reconnaît le principe de sa culpabilité se voit proposer une peine par le procureur de la République. Si elle accepte cette peine, celle-ci devient exécutoire après homologation par un magistrat du siège. Cette procédure, dans laquelle les faits ne sont examinés que de manière très superficielle et dont la publicité est limitée à une fenêtre de quelques minutes au cours de laquelle le fond n'est pas abordé, ne constitue qu'un mode dégradé de gestion productiviste des flux dans un contexte de pénurie de moyens matériels et humains. Le législateur de 2004 avait expressément interdit le recours à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour les délits prévus par des lois spéciales, cette disposition visant à titre principal et spécifique le délit de fraude fiscale. Il avait en effet été considéré avec raison que l'exemplarité attachée aux poursuites pénales de ce chef était incompatible avec une procédure dont les principales caractéristiques sont la superficialité et la discrétion. En application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel précisant les conditions du cumul des sanctions fiscales et des sanctions pénales, la justice ne peut connaître que des faits de fraude fiscale présentant une toute particulière gravité en raison des montants fraudés, du mode opératoire adopté ou de la qualité particulière du fraudeur. dit, s'il existe un domaine du droit où l'on ne peut mettre en oeuvre le plaider-coupable, c'est bien celui de la fraude fiscale ! Quel est l'objectif de l'article 9 ? Dans les faits, essentiellement dispenser un certain nombre de justiciables jouissant d'une assez bonne réputation de se retrouver confrontés aux tourments d'une justice qui viendrait à s'appliquer dans toute sa rigueur et, ne l'oublions pas,

se déroule sous le contrôle d'un juge et permet d'obtenir une condamnation plus rapide. Nous sommes favorables à ce type de procédures qui contribuent à désengorger nos tribunaux correctionnels et qui n'ont, bien sûr, rien d'automatique, puisqu'elles sont proposées

l'impasse sur l'étape de reconnaissance de la culpabilité. Dès lors que cette procédure est ouverte à toute une série d'infractions, il n'y a pas de raison d'en exclure la fraude fiscale. En dépit de

présenter l'amendement n° 85. Nous avons déposé cet amendement de suppression pour avoir un débat sur l'opportunité d'une telle mesure. La commission des lois a adopté un amendement qui autorise la conclusion d'une convention judiciaire d'intérêt public en matière de fraude fiscale. Lors des réflexions préparatoires à la loi du 9 décembre 2016, l'application de cette convention à l'infraction de fraude fiscale a été écartée en raison de son particularisme procédural. Outre le fait que sa philosophie repose sur la prévention et la détection des comportements infractionnels, la convention judiciaire d'intérêt public ne s'applique qu'aux personnes morales. Si cette convention présente un intérêt, la rédaction actuelle n'apporte pas les garanties suffisantes à sa bonne utilisation elle doit être un outil pour renforcer la transparence des comportements et sanctions et doit s'inclure dans une réflexion générale de politique pénale en matière fiscale. De plus, le dispositif proposé pose la question de l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale. La convention La convention judiciaire d'intérêt public est mise en oeuvre si l'action publique n'est pas encore engagée, donc au stade où il est possible pour l'administration de transiger, en application de l'article L.247 du livre des procédures fiscales. Enfin, la lutte contre la fraude fiscale nécessite une validation de la culpabilité. Or la convention judiciaire d'intérêt public n'entraîne pas cette déclaration de culpabilité et n'a pas valeur de jugement. Pour ces raisons, le dispositif tel qu'il est prévu paraît peu opportun.

La CJIP comporte une dimension transactionnelle : il s'agit de trouver un accord plutôt que d'engager des poursuites, moyennant le paiement d'une amende d'intérêt public et la mise en place d'un programme de mise en conformité. Cet outil, vous l'avez rappelé, ma

d'euros. Naturellement, l'opportunité de proposer une CJIP sera appréciée au cas par cas par le parquet dans le cadre de la politique pénale définie par le Gouvernement. tout son sens lorsqu'une entreprise a changé de dirigeants et que la nouvelle équipe a envie de solder le passé en trouvant un accord sur le règlement d'une affaire ancienne de fraude fiscale, tout en mettant en oeuvre un plan de mise en conformité. C'est pourquoi la commission des lois émet un avis défavorable sur ces amendements

Cette convention a pour objet d'imposer à la personne morale mise en cause, en échange du renoncement aux poursuites par le procureur de la République, les obligations suivantes : verser une amende transactionnelle dite d'intérêt public, se soumettre à un plan de prévention de la corruption et réparer les dommages causés par l'infraction. Créée par la loi du 9 décembre 2016, dite loi Sapin II, la convention susdite constitue un mécanisme transactionnel permettant un traitement efficace et rapide des procédures ouvertes pour les faits de corruption, de trafic d'influence et de blanchiment de fraude fiscale, initialement élaboré pour les infractions d'atteinte à la probité. La nouvelle extension aux faits de fraude fiscale emporte deux conséquences. D'une part, elle permet de contourner le verrou, puisqu'il s'agit d'une forme de transaction judiciaire qui ne constitue pas une poursuite. D'autre part, en l'absence de jugement de condamnation, la répression pénale est susceptible de perdre toute sa spécificité, puisqu'elle se rapprocherait du mode de règlement transactionnel effectué par l'administration fiscale. Il pourrait être alors paradoxal de vouloir que l'autorité judiciaire puisse se saisir du dossier de fraude fiscale

et une baisse du chiffre d'affaires des buralistes. Ce n'est pas ce que nous constatons depuis le début de l'année, parce que nous avons beaucoup renforcé les contrôles à la frontière andorrane. Je me suis moi-même rendu en Andorre pendant trois jours, afin de rencontrer le Premier ministre andorran, qui s'est engagé à une diminution de la production

le commerce illégal de cigarettes, en particulier les achats transfrontaliers et je ne peux qu'approuver totalement, sur le fond, les deux amendements qu'a déposés le Gouvernement sur ce sujet.

nuit gravement à la santé publique- ce n'est pas le sujet aujourd'hui -, représente un manque à gagner considérable pour les recettes de l'État et alimente l'économie grise. À l'échelon mondial, la contrebande et la contrefaçon continuent de représenter une perte fiscale de l'ordre de 10 milliards d'euros. En 2017, les services douaniers ont saisi 350 tonnes de tabac de contrebande, un niveau record ayant été atteint en 2015 avec 630 tonnes. L'augmentation des saisies douanières ces dix dernières années confirme qu'une intensification des trafics s'opère. Or plusieurs études ont prouvé que la contrebande de tabac nourrit non seulement la délinquance, mais aussi les mafias, voire le terrorisme. Le rapport de 2015 intitulé, le terrorisme. Le rapport de 2015 intitulé, publié par le Centre d'analyse du terrorisme, démontre que la contrebande de cigarettes représente plus de 20 % des sources criminelles de financement des organisations terroristes,

de la Commission européenne qui dispose : « La contrebande de cigarettes constitue une source de revenus pour les groupes criminels organisés d'Europe. » Enfin, le 26 avril dernier, lors de la Conférence de lutte contre le financement de Daech et d'Al-Qaïda, le commissaire européen au budget lui-même, l'Allemand Günther Oettinger, a indiqué qu'il ne fallait pas seulement limiter la contrebande du tabac aux problématiques de santé publique et de fiscalité, mais qu'il fallait considérer que « la contrebande est devenue une source majeure de revenus pour le crime organisé, et même parfois une source de financement du terrorisme ». Il est donc proposé d'aggraver les peines encourues pour trafic de cigarettes lorsqu'il est commis en bande organisée, et de permettre l'usage de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisée. L'amendement

vous en prie, mon cher collègue. Peut-on examiner un texte relatif à la lutte contre la fraude sans évoquer la lutte contre le trafic de tabac qui entraîne de lourdes pertes fiscales pour l'État et de nombreuses fermetures de bureaux de tabac, commerces de proximité essentiels sur nos territoires ? Lors de la présentation du bilan des douanes, dont je salue ce soir l'action, le travail et les résultats, vous aviez, monsieur le ministre, fait de la lutte contre le trafic de tabac une priorité du quinquennat.

Aujourd'hui, la peine d'emprisonnement est d'une durée de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à dix fois la valeur de l'objet de la fraude lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté ministériel.

Avec le paquet neutre et la hausse du prix du tabac, de plus en plus de Français s'approvisionnent à l'étranger ou sur le marché parallèle, au détriment des buralistes, qui sont très fortement touchés. L'Office européen de lutte antifraude, précise que la contrebande de tabac entraîne chaque année des pertes importantes pour les budgets des États membres de l'Union européenne et de cette dernière, sous la forme de droits de douane et de taxes éludés. Les ventes de tabac de contrebande ne respectent aucune règle et représentent un risque considérable pour les consommateurs et les entreprises. Elles nuisent aux campagnes de santé publique et de lutte contre le tabagisme. De surcroît, elles enfreignent les règles strictes que l'Union européenne et les États membres ont fixées quant à la fabrication, à la distribution et à la vente. Ainsi, la contrebande de cigarettes et des autres produits du tabac est un phénomène mondial, qui, au sein de la seule Union européenne, inflige une perte annuelle de plus de 10 milliards d'euros de recettes fiscales.

amendement a pour objet les dispositifs très ingénieux mis en oeuvre par les trafiquants pour rendre la contrebande et la contrefaçon relativement libres d'accès.

Le marché parallèle sur internet connaît un essor préoccupant, alors même que la loi interdit la vente et l'achat de tabac en ligne. Ainsi, le code général des impôts indique que la vente à distance de produits du tabac manufacturé, y compris lorsque l'acquéreur est situé à l'étranger, est interdite en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Il en est de même de l'acquisition, de l'introduction en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne ou de l'importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d'une vente à distance. Sur le Sur le modèle de la répression des activités illégales de jeux d'argent, cet amendement tend à imposer aux fournisseurs d'accès à internet de prévoir un dispositif informant de l'illégalité et des risques encourus pour l'achat de tabac sur internet.

Ce sujet relève peut-être du domaine des lois de finances ; mais n'est-il pas temps de mettre fin à ce régime dérogatoire accordé à la Corse depuis le Consulat de Napoléon Bonaparte ?

celle des transferts d'actifs à effet retard, si l'on peut dire, à savoir l'ensemble des processus qui, au sein d'un groupe donné à base française et à vocation internationale, peuvent conduire à modifier la domiciliation de certains actifs, dont le potentiel de valeur ajoutée peut venir à manquer au moment d'établir la contribution fiscale de l'entreprise en France. C'est évidemment le cas dès lors que l'on procède à des mouvements sur les éléments matériels du patrimoine de l'entreprise, par exemple, quand on déplace des machines sur un autre lieu de production. Ces

de départ. Combien de nos PME familiales ont connu des fortunes diverses, après avoir été approchées par des investisseurs qui ont récupéré, au fil de leur participation à la transmission de l'entreprise, les meilleurs morceaux

? Il s'agit donc de poser une vraie question, qui va bien au-delà, me semble-t-il, du simple respect de la liberté d'entreprendre. Dans un groupe industriel et commercial donné, dès lors que l'on déplace un brevet, les revenus tirés de l'exploitation de ce brevet se déplacent également ! Quel

sur l'évasion et la fraude fiscales. En s'inspirant de la législation que le Royaume-Uni a adoptée en 2004 et dont l'efficacité préventive a été démontrée, il s'agit de créer, sous peine d'amende, une obligation, à la charge du promoteur du schéma d'optimisation fiscale- il s'agit la plupart du temps d'un cabinet de conseil -ou, à défaut, de son utilisateur, de communiquer le contenu du montage à l'administration fiscale dès les pourparlers de vente de vente ou d'achat du dispositif. Une phase expérimentale pourrait consister à permettre aux cabinets d'avocats ou de conseil qui le souhaitent de communiquer à l'administration les montages dont ils connaissent l'existence, mais qu'ils refusent de mettre en place pour leurs clients.

: La parole est à M. Patrice Joly. Mes chers collègues, cet amendement vise à rénover les critères d'identification des États ou territoires non coopératifs plus communément appelés paradis fiscaux.

l'action menée à ce titre sur quatre critères objectifs. Les trois premiers critères ont été publiés et adoptés par le Conseil de l'Union européenne le 5 décembre dernier. Plus ambitieux, critère permet de sanctionner les régimes fiscaux dommageables. Il repose sur les conclusions du conseil Ecofin du 1 décembre 1997, en matière de politique fiscale. du premier critère, il faut avoir reçu l'évaluation largement conforme du Forum mondial, pour ce qui concerne les échanges d'informations et de données. Le deuxième critère est la participation aux conventions multilatérales ce qui concerne l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Le troisième critère est la mise en oeuvre des mesures minimales anti-BEPS, afin de lutter contre l'érosion des bases fiscales et le transfert de bénéfices.

: avoir un niveau d'imposition inférieur à la moitié du taux effectif moyen de l'Union européenne ; présenter une absence de transparence quant aux structures et aux bénéficiaires effectifs ; réserver des avantages fiscaux à des non-résidents

des paradis fiscaux ; il ne suffit pas de fixer des critères, il convient d'en vérifier l'application. Enfin, une clause de sauvegarde porte sur les pays reconnus comme moins avancés, qui ne disposent pas d'un centre financier : il convient de ne pas les pénaliser.

et d'entreprises à vocation internationale qui n'apprécient guère que leurs activités et placements fassent l'objet d'une trop grande publicité. Cette transparence est un mal nécessaire. Le combat doit être mené ; il est utile pour que les mentalités évoluent au moins autant que les termes de l'échange entre ce que l'on appelle le Sud

européens tels que les Pays-Bas, l'Irlande ou le Luxembourg. Ces juridictions ont en effet été évoquées dans divers scandales au cours de ces dernières années. Si l'Union européenne est elle-même en pointe dans la lutte contre l'évasion fiscale, ce n'est pas le cas de tous ses membres. L'existence de pratiques aussi inventives que le « sandwich hollandais » ou les rescrits accordés aux multinationales, comme à Apple par l'Irlande, le démontrent. Le Parlement européen lui-même, dans son ensemble, a regretté que les États membres de l'Union soient exclus de la liste noire

Rappelons les propos du Président de la République lui-même, dans son discours de la Sorbonne du 26 septembre dernier : « cette divergence fiscale nourrit une forme de désunion, désagrège nos propres modèles et fragilise toute l'Europe [ ...] On ne peut pas bénéficier de la solidarité européenne et jouer contre les autres.

L'article 11 présente quelques défauts, dont le moindre n'est pas de conditionner l'existence d'une liste noire à une forme d'accord européen, puisque la liste produite par le conseil des ministres des finances aurait plus de sens que celle que le travail

et gérés par des États membres de l'Union européenne bénéficient d'une sorte de présomption d'innocence quant au respect des recommandations internationales en matière de transparence fiscale. C'est oublier que l'Europe ne comprend pas que des États et territoires parfaitement coopératifs et libérés de la pression du moins-disant fiscal. L'Europe, c'est, bien sûr, le couple franco-allemand, si souvent célébré, c'est l'Italie, la Pologne, la Slovénie ou la Catalogne, mais c'est aussi Jersey, Guernesey, l'île de Man, l'archipel des Açores, les Canaries, sans parler de Saint-Martin, d'Aruba, de Curaçao, de la Polynésie française, ou encore du Luxembourg, des irlandais et de la discrétion des banques autrichiennes.

à l'échelle planétaire, devant des pays comme le sultanat de Brunei, les Bahamas, mais aussi le Mozambique, la République du Congo ou encore le Tchad, l'Arménie et Madagascar, excusez du peu

une arrière-cour étrangement peuplée, qui mérite, pour le moins, que nous nous y intéressions.

la volonté de la commission et de son excellent rapporteur de favoriser l'échange automatique de renseignements sur les comptes financiers, il n'est pas favorable à l'évolution proposée. D'abord, parce que l'effectivité de l'échange automatique de renseignements est déjà prise en compte par la liste européenne des pays et territoires non coopératifs.

de support juridique permettant l'échange automatique ne signifie pas nécessairement que l'autre État ne coopère pas avec la France. Comme l'a très bien dit M. le sénateur du groupe La République En Marche, il s'agit d'un amendement pragmatique. L'amendement n° 12, présenté par MM. Bocquet,

se fait en appliquant les critères définis à l'article 238-0 A du code général des impôts. Deux éléments sont pris en compte pour décider de l'inscription ou de la radiation d'un État de cette liste, à compter du 1 janvier de l'année l'existence d'un accord fiscal avec la France ou, en l'absence d'un tel accord, la qualité de la coopération fiscale. Nous avons déjà vu quelles évolutions implique cet article du projet de loi, avec la fusion des listes française et européenne. Ainsi, il est prévu de radier les

sont inscrits sur la liste des États et territoires non coopératifs, ou ETNC, ceux qui ont conclu une convention avec la France dont la mise en oeuvre est insatisfaisante ou qui, n'ayant pas signé un tel accord, ont décliné la proposition française ou ont été jugés non coopératifs par le Forum

Durant cette année, les flux financiers vers cet État, peut-être hâtivement radié, pourront échapper aux mesures de rétorsion prises en pareil cas, telles que la majoration des taxations sur de nombreux flux à destination et en provenance des États et territoires concernés. Ce manque à gagner fiscal est regrettable. est regrettable. Pour l'éviter, il conviendrait de revoir les critères de radiation de la liste française des ETNC : un État ne devrait pas être radié de la liste, et donc qualifié de

et référons-nous à la liste établie par le Groupe d'action financière, le GAFI, un organisme adossé à l'OCDE et chargé de promouvoir des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques à l'égard des normes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. On ne peut pas dire que la fraude fiscale soit éloignée de ses compétences, tant elle entre explicitement dans le champ des infractions Il me semble donc que nous pourrions inclure les pays identifiés par le GAFI dans les ETNC français. Cela permettrait de mieux prendre en compte les enjeux de la lutte contre le blanchiment, contre la corruption et contre le financement du terrorisme, dont les liens avec la fraude fiscale internationale sont particulièrement bien documentés.

des normes de l'Organisation de coopération et de développement économiques en matière d'échanges et de renseignements. En l'absence d'évaluation,

vous faites confiance sur parole : alors que l'on connaît très bien les difficultés de contrôle des conventions fiscales internationales et le manque d'effectivité

nombreuses règles de reporting montrent que de grandes banques françaises disposent d'implantations dans des paradis fiscaux. On peut même penser que les vingt plus grandes banques européennes

vise à renforcer la lutte contre les pratiques de certaines banques en matière d'évitement fiscal. Afin de ne pas affecter la conduite d'activités bancaires légitimes dans certains États non coopératifs, comme le financement de projets de développement, l'interdiction est ciblée sur les comportements les plus dommageables. Je pense qu'il est temps d'envoyer un signal clair pour faire en sorte que nos banques ne participent plus, par leur présence et leur implantation sans activités réelles dans des paradis fiscaux, à ces grandes machines à laver de l'argent.

Cet amendement s'inspire d'une proposition de la mission de l'Assemblée nationale relative à la poursuite des infractions fiscales. Cette mission relève que la cellule de renseignement financier nationale apporte une plus-value importante pour la détection des fraudes fiscales qui reposent sur le transfert de fonds vers les paradis fiscaux, ou encore en matière d'organisation d'insolvabilité ». Aujourd'hui, le code monétaire et financier permet à TRACFIN de transmettre à l'administration fiscale des informations sur des faits pouvant relever de la qualification de fraude fiscale ou de blanchiment de fraude fiscale. Selon le rapport Cariou, ce dispositif a permis de procéder à des rappels d'impositions et de pénalités à hauteur de près de 900 millions d'euros. Toutefois, en l'état du droit, la transmission de ces notes au procureur de la République financier n'est pas prévue. Cet amendement

directive anti-blanchiment prévoit la création dans chaque pays de registres publics des sociétés, afin d'identifier les véritables propriétaires et détenteurs d'actifs des structures. des structures. La directive précise que « les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs soient accessibles dans tous les cas » à tout membre du grand public.

telle que l'interdiction des transferts de fonds vers certains pays décidés par l'Agence française de développement, l'AFD. Cette agence a développé un code de conduite dans lequel cette exigence figure. Le présent amendement vise à donner une valeur législative à ce code de conduite.

L'article 12 porte sur une question assez essentielle dans le travail de l'administration fiscale aujourd'hui : celle de l'état des lieux annuel de la pratique de la transaction en procédure contentieuse.

La transaction est fort utilisée en matière de contrôle douanier ; elle est même le mode de résolution par excellence de dossiers de contentieux. Elle est également employée de longue date pour les impôts gérés par la DGFiP. cas notamment parce que chaque dossier d'une certaine importance et concernant des fraudes d'un montant significatif pose la question de la capacité immédiate du contribuable concerné à faire face à ses obligations. En clair, il s'agit de mesurer la capacité contributive du redevable et d'adapter la décision finale à cette capacité. Nul besoin, par exemple, de « charger la barque » lorsque les impôts dus par une entreprise risquent de mettre en péril son existence même, avec la perspective, pour le Trésor public, de se retrouver avec une admission en non-valeur. La transaction peut fort bien consister à prévoir un échéancier de paiement des droits et impôts dus, assortis de pénalités dont le montant pourra éventuellement être réduit à raison des efforts et versements accomplis par le redevable. Sur cet article, nous avons déposé deux amendements, dont l'un soulève, semble-t-il, des questions de constitutionnalité. Posons-nous cependant cette question préalable : l'organisation d'un débat au sein des assemblées sur les questions de recouvrement des créances fiscales impayées et des transactions réalisées dans ce cadre ne pourrait-elle pas faire l'objet d'une modification de la loi organique relative aux lois de finances ou de l'ordonnance relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ?

charge le ministre du budget de publier chaque année un rapport sur l'application de la politique de remises et de transactions à titre gracieux réalisées par l'administration fiscale.

M. Didier Rambaud. L'article 12 prévoit que les transactions d'un montant supérieur à 200 000 euros ou qui portent sur des faits ayant fait l'objet d'une plainte de l'administration fiscale seront notifiées, une fois par an, au président et au rapporteur général des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cette notification mentionnerait « l'identité du contribuable, le montant de l'atténuation accordée et les motifs ayant conduit l'administration à l'accorder. » Notre amendement vise à supprimer cette notification, au motif que la communication de telles informations, notamment

comme de l'Assemblée nationale d'ailleurs, au problème de la procédure pénale en matière fiscale pour trouver un nouvel équilibre entre la toute-puissance des directions de l'administration, y compris à l'encontre, bien souvent, des initiatives mêmes des services déconcentrés, et le pouvoir discrétionnaire de la commission des infractions fiscales, Le Syndicat de la magistrature, dans son mémoire relatif au texte, indique : « Le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude s'inscrit dans une démarche, quasi assumée dans l'exposé des motifs, de compensation de l'indulgence affichée envers les fraudeurs à l'occasion du projet de loi " pour un État au service d'une société de confiance " et du refus déterminé de levée du " verrou de Bercy Le présent projet de loi est néanmoins très modeste dans son ambition, se contentant pour l'essentiel d'aménagements à la marge, de modifications cosmétiques et d'un renforcement des sanctions fiscales administratives qui s'inscrit avant tout dans une volonté de marginaliser la poursuite pénale des auteurs de délits fiscaux, de légitimer le maintien d'un traitement principalement administratif de la fraude fiscale et de tenter de rendre politiquement acceptable la conservation d'un verrou de Bercy, lequel constitue pourtant une spécificité difficilement défendable.

Cela passe par la rupture claire avec la logique de suppression massive de postes de fonctionnaires au sein des administrations fiscales qui a sensiblement appauvri la qualité du travail accompli, malgré le profond sens de l'intérêt général qui anime leurs 125 000 agents. Il convient de lancer le service public fiscal à la reconquête de ses positions perdues pour donner une inflexion réelle à la lutte contre la fraude sociale, comme fiscale, et résoudre, en connaissance de cause, la fameuse dialectique du verrou de Bercy. Plus de moyens matériels et humains, une étude conjointe de l'administration et de la juridiction compétente des dossiers nécessitant une procédure judiciaire, voilà comment sortir des controverses actuelles par le haut. L'intérêt général ne le vaut-il pas ?

aujourd'hui, tel qu'il est rédigé, le texte ne supprime pas le verrou de Bercy, puisque le dispositif proposé s'ajoute à la règle inscrite du verrou de Bercy ; il ne s'y substitue pas. Cela a pour conséquence extrêmement simple que le juge ne peut se saisir, sans l'avis du ministère de l'économie

sont donc définis pour être applicables sans obligation de cumul entre eux. Voilà qui permettra, à notre sens, de sortir- enfin ! -du verrou de Bercy, qui crée, par son opacité,

monsieur le ministre.

Monsieur le ministre, le procureur n'a pas de don de divination. Si l'administration fiscale ne lui transmet pas les dossiers, ne lui précise pas que tel ou tel fait l'objet d'une enquête,

Le scrutin est ouvert.

que le régime applicable aux poursuites concernant une autre infraction, en l'occurrence la fraude fiscale, ne lui est pas applicable. Ensuite, le souci de lisibilité milite pour que les dispositions procédurales permettant la répression des infractions prévues par le code pénal

inscrire la jurisprudence dans la loi, afin de sécuriser les procédures engagées sur ce fondement, ces procédures pouvant être mises en cause à n'importe quel moment si un revirement de jurisprudence intervenait. Pour justifier la suppression de cette disposition, le Gouvernement avance des arguments de forme, dont aucun ne nous paraît vraiment décisif. Bien sûr, il est sans doute possible d'affiner davantage la rédaction de cet article, et nous serons ouverts aux améliorations

le champ d'application de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, lequel ne s'applique aujourd'hui qu'à la fraude fiscale et non au blanchiment de ce délit. Ce point a été longtemps discuté avant d'être tranché par l'arrêt de la Cour de cassation en 2008 qui permet au parquet de s'autosaisir des cas de blanchiment. Il n'est donc pas inutile que le législateur confirme cette solution jurisprudentielle, afin que l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre la fraude fiscale travaillent dans un environnement juridique sécurisé.

Cet amendement vise à modifier la définition de l'abus de droit, dispositif qui permet à l'administration fiscale de sanctionner les pratiques d'optimisation abusive. En effet, l'article L. 64 du livre des procédures fiscales permet à l'administration fiscale d'écarter, pour l'établissement de l'impôt, les actes constitutifs d'un abus de droit, définis par deux critères alternatifs : soit les actes en cause sont fictifs, soit ils méconnaissent l'esprit de la loi, dans le but exclusif d'échapper à l'impôt. Ainsi, la faiblesse essentielle de l'abus de droit est d'être assez aisément contournable par la mise en avant d'un élément économique, même très ténu. En 2013, le président de la commission des finances du Sénat de l'époque, Philippe Marini, a déposé une proposition de loi visant à modifier cette définition, en précisant que les actes en cause pouvaient avoir pour motif essentiel et non exclusif d'échapper à l'impôt.

suite du rapport rendu par l'ancien député Pierre-Alain Muet, c'est finalement le terme « principal » qui a été choisi. La nouvelle définition a été adoptée définitivement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014. cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel, ce que l'on peut très fortement regretter. Cet amendement a pour objet de relancer le débat sur l'abus de droit,

nous ne pouvons évidemment pas apporter notre soutien à ce texte, qui, au regard des enjeux, nous semble

que ce problème méritait bien davantage ... Nous enregistrons un certain nombre d'avancées : c'est évident. Cependant, la déception est grande, notamment à propos du verrou de Bercy

La lutte contre la fraude fiscale doit rester une priorité, à la fois parce que le consentement à l'impôt repose sur le fait que tous ceux qui ne s'y soumettent pas doivent être poursuivis

il n'y a jamais eu autant d'argent sale dans les paradis fiscaux, avec des systèmes de plus en plus sophistiqués. Quelques pays continuent à jouer l'opacité, sans être forcément étiquetés comme des paradis fiscaux. Prenez Dubaï, qui n'est pas sur notre liste : ils n'exécutent pas les mandats d'arrêt et ne coopèrent pas. Si je suis un fraudeur, je vais y mettre mon argent ». Mais il ne faut pas se faire d'illusion, les temps changent très vite ! Nous nous inscrivons dans ce mouvement, patient,

collaborative au niveau d'internet. Il y a encore du chemin à faire, mais il faut avancer pas à pas. Nous pensons également qu'il faudra, en corollaire, continuer à simplifier

de la commission des finances et celle de la commission des lois, nonobstant ce que j'ai entendu. Il s'agit de quelques scories qui sont tout à fait dommageables. Malgré cela et bien